monsieur le président.

L'ordre du jour appelle la désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur la souveraineté numérique, créée sur l'initiative du groupe Les Républicains en application du droit de tirage prévu par l'article 6 du règlement.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 heure. Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement.

résolument engagée en faveur de la biodiversité. Je salue cette marque d'engagement, qui s'accélère fortement depuis la création de l'Agence française pour la biodiversité en 2017. L'article 1 de ce projet de loi crée l'Office français de la biodiversité, reprenant les missions de l'AFB et de l'ONCFS, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. exercera ainsi la police administrative et judiciaire relative à la chasse et à la pêche, afin de mieux la répartir dans l'espace et dans le temps. Davantage d'efficacité est ainsi attendue sur le terrain.

réel équilibre entre les chasseurs, les pêcheurs, les forestiers, les agriculteurs et les associations environnementales. Enfin, j'appelle votre attention sur la boulimie ou la frénésie législative en matière de politique environnementale.

et, en bonne fée, de lui donner toutes ses chances, en le parant de dons propres à lui garantir un avenir, sinon radieux, du moins stable et prometteur. La loi de 1976, ambitieuse et sans précédent, instaurait un « un « patrimoine naturel d'intérêt général ». Dans la lignée de cet héritage, je propose de nommer cette nouvelle instance « Office français de la nature », une dénomination susceptible d'englober tous les sujets concernés, non seulement la chasse, mais aussi la pêche, les paysages et les écosystèmes.

du code de l'environnement : « On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants. » Ces interactions peuvent bien évidemment être positives ou négatives. Il nous semble donc que la biodiversité

En isolant la chasse, on donne l'impression qu'elle n'a pas de lien avec la biodiversité et qu'on cherche à la séparer des enjeux de préservation de la biodiversité. Même si tel n'était pas l'objectif de la commission, le résultat masque, de fait, les autres missions de la nouvelle agence. agence. Si l'on tient vraiment à ce que la chasse apparaisse dans le nom, il conviendrait de lister tous les usages de la biodiversité. Cet organisme devrait donc s'appeler Office français de la biodiversité, de la chasse, de la pêche, de la cueillette, du pastoralisme, etc. Je suis volontairement

sur ces amendements, qui visent à revenir sur la position de la commission. Nous avons tenu à ce que l'Office français de la biodiversité soit renommé « Office français de la biodiversité et de la chasse Il nous paraît particulièrement important d'ouvrir nos débats en rappelant notre souci de préserver l'identité des deux entités fusionnées, afin que l'une ne se sente pas absorbée par l'autre.

et celle de Mme la rapporteure pour avis de la commission des affaires économiques. La fusion de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage doit doit se faire dans le respect de chacun. Or, madame la secrétaire d'État, quinze jours après l'adoption du texte en conseil des ministres, vous déposiez un amendement en commission à l'Assemblée nationale sonnant la fin de la concertation et imposant le nom « Office français de la biodiversité

Mes chers collègues, je vais vous raconter une histoire de nature. Sur les hauts plateaux du Vercors, où le sol est constitué de calcaire poreux, l'eau est rare. Il a été observé que le cerf y aménage des baignoires imperméables, en se roulant dans la boue. Grâce à des photos prises par des naturalistes, on a pu constater que ces souilles servent d'abreuvoirs à d'autres animaux, comme le chevreuil, la martre, le lièvre, voire le loup.

Le scrutin est ouvert.

Le présent amendement introduit la notion de « protection des espèces », qui est plus large que celle de « surveillance, préservation, gestion et restauration de la biodiversité

Permettez-moi, avant toute chose, d'indiquer que le texte initial, qui ne comprenait que six grandes catégories de missions, a été substantiellement enrichi par nos collègues de l'Assemblée nationale, qui ont porté ce nombre à Bien que je ne nie pas l'intérêt qu'il y a à préciser le champ d'action d'un établissement public d'une telle importance, je souhaite souligner que, le nouvel établissement disposant à peu près des mêmes ressources, à quelques dizaines de millions d'euros près, que les deux établissements qu'il entend rapprocher, il me paraît dangereux d'élargir ce périmètre outre mesure et de pécher par excès d'ambition. C'est pourquoi la commission vous proposera de rejeter les extensions de périmètre qui semblent déjà satisfaites par la lettre du texte actuel ou qui se contenteraient de retranscrire de grands principes dans un article à vocation essentiellement opérationnelle. En l'espèce,

Biodiversité et stabilité climatique sont étroitement liées. Le besoin de coordination est réel, comme en témoigne le besoin, notamment exprimé par les acteurs du monde agricole, de penser les politiques de l'eau en lien étroit avec celles d'adaptation au changement climatique, et cela dans un contexte où les activités agricoles sont elles-mêmes appelées à participer à l'effort de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il est impératif de penser la protection de la biodiversité en lien avec la lutte contre le changement climatique afin d'éviter la mise en place de mesures favorisant l'une, mais nuisant à l'objectif global de préservation de conditions de vie et de développement soutenables à long terme.

En effet, elle s'est prononcée en faveur d'un rehaussement de la mission de police dans l'énumération des missions du futur établissement. Cette mesure, quoique dépourvue d'effets juridiques, n'est pas uniquement symbolique. Elle rappelle utilement que les agents chargés de la mise en oeuvre de la politique de la biodiversité sont investis d'une mission avant tout régalienne. À mon sens, la lutte pour la préservation de l'environnement passe aussi par la réaffirmation de ce principe. Quel est l'avis du Gouvernement

Enfin, comme cela a été souligné lors des débats à l'Assemblée nationale, le développement durable de la chasse relève des fédérations des chasseurs, et non de l'OFB. Les

au sein des parcs animaliers, tel celui du Gévaudan. Devant la recrudescence des attaques, notamment contre les troupeaux, il importe que les agents de la nouvelle entité s'assurent que les loups qui évoluent en semi-liberté restent à l'intérieur du périmètre clôturé. Je précise que cette mission d'observation doit s'effectuer à moyens constants.

deuxième domaine maritime mondial, la France héberge 10 % de la biodiversité de la planète, dont la majeure partie en outre-mer.

C'est dire l'importance scientifique que présentent ces régions, dont certaines spécificités sont peu ou mal prises en compte au niveau national. Ainsi, selon le rapport de 2018 de l'AFB, la biodiversité ultramarine, qui se caractérise

les espèces exotiques envahissantes menacent l'équilibre des écosystèmes indigènes. Elles entrent en concurrence directe avec les espèces autochtones. Selon l'Union internationale pour la conservation de la nature, elles constituent l'une des premières causes d'érosion de la diversité biologique au niveau mondial, après la disparition et la fragmentation des habitats.

Bien que l'éradication des espèces envahissantes soit difficile, des actions de prévention et de limitation peuvent être envisagées et mises en oeuvre. L'inventaire de ces espèces et l'étude de leur dynamique

de 2018, seulement 29 % des grands groupes taxonomiques bénéficiaient d'un référentiel satisfaisant au regard des connaissances disponibles dans les territoires ultramarins, avec de fortes disparités

s'agissant des collectivités d'outre-mer frontalières d'autres États avec lesquels elles partagent des problématiques territoriales similaires en termes de maintien de la biodiversité et de lutte contre la pollution,

Or les collectivités d'outre-mer abritent près de 10 % des récifs coralliens existant dans le monde, ce qui justifie une action de protection des coraux et de surveillance particulière dans ces territoires. L'initiative française pour les récifs coralliens, l'Ifrecor, a précisément été lancée en 1999 à cette fin. Sa mission est la gestion durable des coraux des collectivités françaises d'outre-mer et de leurs écosystèmes associés, tels que les mangroves et herbiers. Dans un souci de cohérence et d'efficacité de la protection des récifs coralliens sur ces territoires, il s'agit d'affirmer le principe de la coopération entre la future OFB et l'Ifrecor. Menacés d'érosion accélérée à l'heure du changement climatique, les coraux sont des animaux essentiels à l'équilibre biologique des milieux marins, et donc au maintien de la biodiversité aquatique. La protection que leur offre l'Ifrecor légitime l'appui de l'OFB dans la réalisation de ses missions.

de la biodiversité porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises. ...] Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie et dans ses provinces, à la demande de ces collectivités. » Le texte a donc explicitement prévu l'intervention de l'établissement dans chacun des territoires ultramarins, compte tenu de leur spécificité juridique.

l'alinéa 19 prévoit que celui-ci devra apporter un appui aux acteurs socio-économiques dans leurs actions en faveur de la biodiversité. Cet amendement vise à étendre cette possibilité de soutien aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, qui sont des acteurs incontournables de la promotion de la biodiversité

L'alinéa 19 prévoit en effet un appui global aux acteurs socio-économiques, et l'alinéa 23 l'accompagnement de la mobilisation citoyenne de la société civile et des acteurs des secteurs économiques pour les enjeux de la biodiversité, notamment le lien entre l'homme et la nature. L'avis est donc défavorable.

appui à l'État et à ses établissements publics [ ...], notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes ». Ce point figure donc déjà dans le texte.

à assurer la sensibilisation à la nécessité de préserver et de reconquérir la biodiversité la formation du plus grand nombre, ainsi qu'à structurer, pour mieux les professionnaliser, les filières de métiers liés à la biodiversité et aux services écosystémiques. Cette sensibilisation doit faciliter la prise de conscience de la responsabilité de tous dans la protection de la biodiversité, contribuant ainsi à créer les conditions d'un engagement progressif de chacun à changer ses pratiques et à agir pour relever ce défi de la reconquête. Elle doit également jouer un rôle primordial en matière d'information sur le fonctionnement des écosystèmes et de prévention des atteintes à la réglementation, qui sont préjudiciables à l'ensemble de la société. Quel

en fonction de la présence territoriale du loup et des dégâts occasionnés. Cela permettrait de répondre concrètement aux attentes des éleveurs, qui n'auraient ainsi pas à attendre l'extension du plan quinquennal précédent. En effet, le plan quinquennal 2018-2023, 2018-2023, publié en février 2018, a particulièrement déçu les élus, les éleveurs et les agriculteurs, qui s'attendaient à davantage de cohérence, alors que le Président de la République avait indiqué

Une collaboration nous permettrait, dans le respect des prérogatives des uns et des autres, de mettre en cohérence les politiques de l'État, de l'OFB et de la collectivité de Saint-Martin. Nous accomplirions ainsi ensemble une mission de pédagogie envers nos populations, permettant d'éviter des tensions, des crispations et des conflits inutiles.

nous ont fait part de la préoccupation légitime de conserver les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Saint-Martin dans le champ conventionnel de l'OFBC. Il est toutefois important de préciser que la signature de conventions

du Gouvernement ? J'ai le même avis que la commission, essentiellement pour les mêmes raisons. Je voudrais confirmer que la convention-cadre qui a été signée en novembre 2018 entre l'État,

Simplement, à côté des activités partenariales, les missions régaliennes de police doivent demeurer dans les mains de l'établissement public. Le même raisonnement s'applique à Saint-Martin. Je mets aux voix le

des activités régaliennes. Il me semble important que cet établissement soit géré dans des conditions qui donnent la majorité à l'État. Néanmoins, compte tenu des questions posées par la taille du conseil d'administration, que nous souhaitons tous raisonnable-

parole est à M. Guillaume Gontard. La gouvernance de ce nouvel opérateur a fait l'objet d'intenses débats, relatifs notamment au nombre d'administrateurs.

Toutefois, comme cela a été rappelé lors des débats à l'Assemblée nationale, le futur office sera un établissement public administratif, dont les prérogatives de police, et donc le caractère régalien, seront particulièrement renforcées, ce qui justifie une représentation majoritaire de l'État. De plus, cette majorité représentera les collectivités territoriales, notamment les outre-mer, qui abritent 80 % de la biodiversité française, mais aussi les établissements publics ayant un rapport avec l'office- cela peut être le cas de l'ONF, par exemple. ailleurs, l'office est non pas un outil de décentralisation, mais un outil national avec des déclinaisons régionales, destiné à assurer la préservation de la biodiversité sur l'ensemble du territoire national. Enfin, nous ne pensons pas que le conseil d'administration puisse être la somme des représentants d'intérêts particuliers. En ce sens, réserver une majorité réservée à l'État garantit aussi une meilleure prise en compte de l'intérêt général.

parole est à M. Daniel Gremillet. Compte tenu du contexte et surtout de la dimension territoriale, nous proposons de prévoir une représentation suffisante, au sein du conseil d'administration, du deuxième collège, qui comprendra « des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et et forestières, d'associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement, des gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir », et de donner ainsi à toutes ces parties, premiers acteurs de la préservation et de la valorisation de la biodiversité, leur juste place au sein de l'établissement.

dont les intérêts sont le plus directement impactés. Il nous semble que c'est ainsi que nous les ferons efficacement participer à la mise en oeuvre des politiques de préservation de la biodiversité. En conséquence, la commission a donné un avis défavorable à l'amendement du Gouvernement,

En cas d'impossibilité d'atteindre un consensus, nous considérons que, compte tenu de la nature de l'établissement, de ses missions de police, de ses pouvoirs régaliens

J'entends bien que la composition par collèges n'a d'incidence que sur la désignation des membres du conseil d'administration, mais il ne serait pas opportun que la loi suggère que leur intérêt à agir soit d'une nature différente de celle des autres acteurs socio-économiques. La commission a donc émis un avis défavorable.

Cette appellation trop générale ne correspond pas à la réalité, une seule structure nationale représentative étant clairement identifiée. La Fédération nationale des chasseurs est composée des fédérations départementales et interdépartementales des chasseurs, et il est donc pertinent de ne mentionner dans le texte que la Fédération nationale Cet amendement de précision est nécessaire pour éviter, à l'avenir, toute difficulté ayant trait à la désignation des représentants de cette fédération nationale, à la fois agréée et parfaitement représentative des activités cynégétiques.

peut-être aussi en qualité

La justification de cet amendement tient au fait que les chasseurs continueront de financer l'établissement, au travers de la redevance cynégétique, à hauteur de 45 millions d'euros, tandis que les pêcheurs contribueront de leur côté pour environ 10 millions d'euros. Les structures de la chasse et de la pêche seront ainsi les seuls financeurs privés du nouvel établissement.

La commission a initialement choisi de fixer un quantum minimal pour la seule représentation des chasseurs et des pêcheurs. Nous avons motivé ce choix par la structuration

Entendons-nous bien, il s'agit non pas d'un traitement de faveur, mais d'un traitement spécifique, qu'appelle la spécificité de leur organisation. Après réflexion, il nous a paru logique que cette spécificité soit étendue aux organisations agricoles et forestières, qui ne bénéficient souvent pas de l'efficacité des têtes de réseau des associations de protection de la nature. Plus que des promotrices de positions unifiées et structurées, elles sont les porte-voix de la pluralité

notamment en matière de réseaux d'eau et d'assainissement. locale de l'eau du risque d'un affaiblissement supplémentaire dont les effets seraient particulièrement dommageables pour les collectivités locales.

des investissements des collectivités territoriales en faveur des réseaux d'eau et d'assainissement. Le principe selon lequel l'eau paie l'eau doit être sacralisé, d'autant que les agences de l'eau

d'économie de la ressource en eau et de recherche de solutions fondées sur la nature. L'ONCFS, en revanche, n'est pas financée par les agences de l'eau. La fusion des deux établissements n'a pas vocation à se traduire par une ponction supplémentaire sur les budgets de

dixième programme était plus élevé, mais ce programme finançait de manière exceptionnelle la mise aux normes d'un certain nombre de stations d'épuration. À l'intérieur du onzième programme, 3,5 milliards d'euros sont affectés directement à l'eau et à l'assainissement. Je confirme,

Estrosi Sassone. Cet amendement vise à demander au Gouvernement de remettre au Parlement, avant le 1 janvier 2020, un rapport sur la méthodologie de recensement et de comptage des loups. Ce rapport pourra émettre des propositions de nature à permettre, le cas échéant, de remédier aux difficultés constatées. Tout le monde s'accorde à reconnaître que la réalité de terrain ne correspond pas du tout

L'État a amorcé, voilà plus de dix ans, l'inventaire national du patrimoine géologique. Le présent amendement vise à la prise en compte, dans le cadre d'une stratégie nationale en faveur de la conservation du patrimoine naturel, des résultats de cet inventaire et de tout autre inventaire géologique à venir soutenu par l'État.

La conservation et la valorisation du patrimoine géologique sont déjà assurées par deux organes particuliers, le Muséum national d'histoire naturelle et le Bureau de recherches géologiques et minières.

Il ne nous paraît pas souhaitable d'élargir son champ au-delà des obligations internationales ni d'ajouter une obligation juridique aux stratégies régionales pour la biodiversité, comme le prévoit le deuxième point de cet amendement. Nous avons déjà intégré la géodiversité en complément de la définition de la biodiversité dans le code de l'environnement.

la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, avec sa formation spécialisée dans l'indemnisation des dégâts de gibier, et la commission départementale

existantes. Quel est l'avis de la commission ? L'évolution proposée par notre collègue ferait perdre aux commissions départementales de la nature, des sites et des paysages leur composante « nature », qui constitue un élément utile à l'appréciation des questions paysagères et patrimoniales. Il nous semble par ailleurs que les évolutions récentes de la gouvernance territoriale en matière de biodiversité conduisent à privilégier l'échelon régional, ce qui ne plaide pas en faveur de la mise en place d'un nouvel échelon départemental. Enfin, il ne nous paraît pas opportun de remettre en cause l'objet actuel et l'existence des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, dont les missions portent majoritairement sur les questions cynégétiques et qui constituent des instances de consultation bien identifiées dans les territoires. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable

principes et règles d'accès, de diffusion et de réutilisation des données publiques qui prévalent aujourd'hui sont définis dans la loi. L'amendement n° 44 Il est essentiel de prévoir que le décret d'application de l'article L. 414-10 devra préciser les missions d'intérêt général assurées par les conservatoires botaniques nationaux, pour mieux les distinguer des activités qu'ils peuvent avoir par ailleurs dans le champ concurrentiel. Ces trois amendements peuvent sembler un peu techniques et guère

rôle majeur, tant pour la connaissance des milieux naturels et des écosystèmes que pour la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la préservation de la biodiversité et à la protection du patrimoine naturel. du patrimoine naturel. Une extension du périmètre de leur action à des pouvoirs coercitifs ne semble pas de nature à assurer une meilleure mise en oeuvre de la police environnementale dans les territoires. Au contraire, le maintien de la distinction entre les volets prévention et répression apporte davantage de garanties en vue d'une meilleure efficacité dans la constatation et la recherche des infractions.

La commission est défavorable à la suppression de cet article, qui étoffe substantiellement les pouvoirs de police judiciaire des inspecteurs de l'environnement. Elle y a apporté plusieurs ajouts, sur lesquels j'aurai l'occasion de revenir. Nous ne sommes

de véhicules, est aujourd'hui restrictif. Il ne concerne en effet que les « véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs utilisés à titre professionnel Or, en matière environnementale, les infractions peuvent être commises avec tout type de véhicules, y compris non professionnels. C'est notamment le cas en matière de chasse et, surtout, d'espèces protégées.

ces deux amendements vont manifestement à l'encontre de ce que l'ensemble des acteurs concernés ont jugé comme une évolution positive, à savoir l'unification des compétences de police environnementale de l'ensemble des polices spécialisées autour d'un socle commun d'infractions. l'efficacité de leur action, la commission a jugé tout à fait opportun d'habiliter les inspecteurs de l'environnement affectés à l'OFBC, où seront représentées l'ensemble des parties intéressées, dont les organisations forestières, à connaître de l'ensemble des infractions, y compris forestières.

les pouvoirs que le texte leur attribue lorsqu'ils agissent en qualité de délégués du procureur de la République, à savoir la possibilité de transmettre une composition pénale et de notifier une convocation en justice. Il a pourtant semblé à la commission que l'explicitation de ces pouvoirs permettrait à la police de l'environnement d'être plus efficace, plus rapide et plus proche des individus sur lesquels elle exerce ses prérogatives. Ces pouvoirs permettront notamment aux

Delattre. En commission, monsieur le rapporteur, vous avez rejeté cet amendement au motif que les gardes particuliers n'auraient pas de prérogatives de puissance publique. Cela n'est pas exact : je vous invite à consulter la convention de partenariat signée en 2016 entre le ministère de l'intérieur et le président de la confédération française des gardes particuliers assermentés, qui précise ces prérogatives. Cet amendement vise à soutenir la lutte contre les atteintes à la biodiversité en coordonnant l'ensemble des ressources à disposition en matière de police environnementale, afin de rendre immédiatement l'organisation de la police judiciaire de l'environnement, et partant le rôle des agents et gardes autres que ceux qui relèvent de l'inspection de l'environnement ou des forces de police générale. Les gardes particuliers sont des acteurs essentiels de la surveillance et de la police rurale de proximité.

des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement avait exclu les gardes particuliers, gardes-chasse, gardes-pêche, gardes-bois, des acteurs de la police de l'environnement. Cet amendement vise donc à remédier à cette maladresse. Quel

habilités à constater des infractions au code de l'environnement dans le strict périmètre des domaines sur lesquels leur assermentation leur confère cette habilitation les pouvoirs d'investigation propres aux inspecteurs de l'environnement, qui sont des agents de droit public et qui disposent d'une compétence de police générale, avec une possibilité d'extension territoriale.

à Mme Sylviane Noël. Pour lutter efficacement contre les trafics de faune ou de flore, les contrôles des moyens de transport sont très efficaces. Cet amendement vise donc à préciser le texte en matière de recherche et de constatation des infractions dans les véhicules et à prévoir la possibilité d'avoir recours à des moyens appropriés pour stopper des véhicules

aujourd'hui réservés aux officiers de police judiciaire chargés de lutter contre les délits de fuite, notamment les dispositifs de type « hérisson ». Compte tenu des pouvoirs de police judiciaire attribués aux inspecteurs de l'environnement, la portée de cet amendement a paru excessive à la commission. Avis défavorable.

des agents de police environnementale. Nous nous sommes montrés attentifs à ce que leurs pouvoirs coercitifs soient utilement réaffirmés, sans pour autant entretenir de confusion dommageable entre les agents de police environnementale et les officiers de police judiciaire. Je rappelle en effet que ces derniers reçoivent une formation spécifique et disposent de locaux particuliers, nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, qui supposent souvent des privations ponctuelles de liberté.